comités exécutifs des entreprises. Il est satisfait : les « instances dirigeantes » visées à l'article 7 incluent bien ces deux instances, dont la définition est par ailleurs introduite dans le code de commerce par la présente proposition de loi.

instance mise en place au sein de la société [ ...] aux fins d'assister régulièrement les organes chargés de la direction générale dans l'exercice de leurs missions ». Le champ d'application de la mesure permet donc bien de viser les membres des comex et des codir. Votre amendement étant satisfait, j'en demande le retrait ; à défaut, l'avis sera défavorable.

est à Mme la ministre déléguée. Le présent amendement vise à clarifier l'appréciation du seuil de 1 000 salariés qui délimite le champ d'application de l'article 7. Doivent être soumises à l'obligation de quotas les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen de plus de 1 000 salariés. d'éviter, par cette précision, qu'une société franchissant ce seuil de façon temporaire ne sache pas si elle doit ou non se conformer aux obligations figurant à l'article 7.

L'objet du présent amendement est d'étendre les objectifs paritaires aux instances de gouvernance de toutes les entreprises d'au moins 250 salariés et présentant un minimum de 50 millions de chiffre d'affaires.

Il est important de noter, comme vient de le faire Mme la rapporteure, que les instances dirigeantes, telles que les comités exécutifs, sont principalement mises en place dans les grandes entreprises. Les cadres dirigeants sont moins, voire très peu, présents dans les entreprises de 250 à 1 000 salariés. Le calcul des écarts de représentation femmes-hommes dans cette population ne serait donc pas pertinent statistiquement. Pour ce qui concerne la condition liée au chiffre d'affaires, les obligations imposées aux entreprises sont traditionnellement fixées dans le code du travail en fonction de seuils d'effectifs qui sont bien connus par les entreprises. Notre objectif est de viser les entreprises ayant une taille assez importante pour être dotées de comités de direction et d'un nombre suffisant de cadres dirigeants. Faire reposer la mesure sur le montant du chiffre d'affaires de l'entreprise rendrait plus complexe la lisibilité du champ d'application de la mesure, mais aussi les contrôles que l'inspection du travail pourrait effectuer. Pour toutes ces raisons, je suis défavorable à ces amendements.

comprenant les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes. Cette notion nous paraît contre-productive, car elle risquerait de limiter la portée de la mesure prévue. En effet, la publication devrait concerner deux deux populations distinctes, d'une part, les membres des instances dirigeantes, et, d'autre part, les cadres dirigeants. Cette précision est importante en vue de renforcer la parité au sein de ces deux sphères permettre à davantage de femmes de prendre part aux instances dirigeantes, et permettre à davantage de femmes d'être cadres dirigeantes. Les chiffres sont là, nous les avons rappelés. Il est donc essentiel d'agir pour que la parité soit assurée partout. Quel est l'avis de

que la publication concerne deux populations distinctes : d'une part, les membres des instances dirigeantes, et, d'autre part, les cadres dirigeants. Elle permet d'éviter l'interprétation selon laquelle un taux de représentativité unique serait calculé en assimilant totalement les cadres dirigeants

la publication des écarts avant cette échéance prévue par l'Assemblée nationale a toute son utilité. Elle permettra de visibiliser « au fil de l'eau » les efforts opérés par les entreprises afin de féminiser leurs instances dirigeantes, et de constituer à la fois une base de données utile

et les hommes soient rendus publics sur le site du ministère du travail un an après l'entrée en vigueur de la loi, et non pas cinq ans après, comme le préconise la commission des affaires sociales. L'article 7 vise à ce que les entreprises parviennent, d'ici dix ans, à déconstruire le plafond de verre dont nous avons hérité, en s'appuyant sur des jalons qui sont autant d'étapes pour atteindre cet objectif. Or décaler un jalon pour le faire concorder avec un autre risquerait de déséquilibrer la progressivité de la méthode proposée à l'article 7. L'obligation de publication ne doit pas être vue, par ailleurs, comme une sanction, mais plutôt comme un outil mis à la disposition des entreprises pour mettre en valeur les efforts consentis et pour attirer les talents. Je pense en particulier aux filières qui peinent à recruter en raison d'un marché des compétences tendu, et qui auront une nouvelle corde à leur arc pour séduire un public qu'elles n'attiraient pas auparavant. Enfin, presque quarante ans après les premiers textes sur l'égalité professionnelle et dix ans après la loi Copé-Zimmermann, on peut raisonnablement penser que les entreprises ont eu largement le temps de s'adapter à cet objectif, et qu'elles peuvent accélérer sans plus attendre cette démarche.

est perçue par les entreprises comme une sanction qui intervient avant l'entrée en vigueur de la loi.

C'est la raison pour laquelle la commission n'est pas revenue sur un autre dispositif de publicité, à savoir la publication des écarts d'égalité hommes-femmes sur le site

de la publication des résultats sur le site internet du ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion le 1 mars de la cinquième année suivant la publication de la présente loi. Ces amendements visent à prévoir, quant à eux, une entrée en vigueur de cette mesure le 1 mars de l'année suivant la publication de la présente loi, conformément au loi, conformément au vote de l'Assemblée nationale. J'entends les arguments de votre rapporteure, qui souhaite laisser plus de temps aux entreprises pour adapter leurs pratiques à la nouvelle réglementation. dans le même temps que, depuis dix ans, les entreprises ont eu suffisamment de temps pour féminiser leurs équipes. Il s'agit ici d'une mesure peu coercitive, qui permettra de recruter sur des secteurs d'emplois aujourd'hui déjà en tension. Il nous faut donc pouvoir définir une entrée en vigueur permettant de concilier l'exigence de transparence, tout en accordant aux entreprises un délai avant que leurs résultats ne soient mis en ligne sur le site du ministère chargé de l'emploi. Ce délai doit permettre aux entreprises de mener les premières actions pour améliorer la parité entre les femmes et les hommes au sein de la population visée. La définition du délai d'entrée en vigueur le plus adéquat pourra faire l'objet d'un compromis dans la suite de la navette parlementaire. Une durée de deux ans avant la publication pourrait, par exemple, être une échéance tout à fait adaptée.

ont employé un nombre moyen de plus de 1 000 salariés. En apportant cette précision, il s'agit d'éviter qu'une société qui franchirait ce seuil de façon temporaire ne sache pas si elle doit se conformer ou non aux obligations figurant à l'article 7. Cette formulation reprend

facultatif de la sanction en renforçant la portée de l'obligation paritaire et en diminuant de moitié le délai de mise en conformité à l'expiration du délai légal. Quel est l'avis de

préciser que l'autorité administrative prend en compte la situation initiale de l'entreprise, les efforts constatés ainsi que les motifs de sa défaillance si elle n'est pas en mesure de satisfaire aux quotas prévus par la loi.

à ajouter un caractère systématique à la sanction en cas de non-atteinte de l'objectif fixé. Le dispositif instauré à l'article 7 fixe des objectifs ambitieux, tout en laissant le temps nécessaire aux entreprises présentant une faible mixité femmes-hommes d'agir sur le vivier de cadres. Soyons réalistes : certaines entreprises partent de si loin et connaissent un niveau de mixité femmes-hommes tellement bas que, pour atteindre les paliers intermédiaires de 30 %

l'inspection du travail doit disposer d'une marge d'appréciation s'agissant de l'application de la sanction afin de pouvoir tenir compte des situations spécifiques des entreprises, qu'il s'agisse des efforts qu'elles vont entreprendre en matière d'égalité femmes-hommes, de leur situation initiale en matière de parité, de parité, du bassin d'emploi, des difficultés économiques éventuelles, etc. Il est donc nécessaire de maintenir le caractère non systématique de l'application de la pénalité. C'est la raison pour laquelle je suis défavorable à cet amendement.

C'est pourquoi le dispositif prévoit une pénalité financière pour l'entreprise, qui ne pourra pas excéder 1 % des rémunérations et des gains versés aux travailleurs salariés au cours de l'année civile précédente.

C'est pourquoi nous proposons d'instaurer un plancher fixé à 0,5 % des rémunérations et gains versés aux travailleurs salariés. Quel

que pas de sanction du tout. Si une entreprise ne répondait pas aux obligations fixées par la loi et que l'administration avait en tête un plancher, tel que

à Mme Laurence Cohen. Nous proposons d'augmenter la pénalité financière prévue au bout de deux ans lorsque les entreprises n'auront pas respecté le quota à atteindre en termes de parité dans toutes les instances dirigeantes. Au-delà du délai de mise en conformité et du seuil à atteindre, sur lesquels il faut être plus exigeant et ambitieux, nous pensons qu'il faut également jouer sur le levier de la pénalité financière. On l'a vu, et cela fait des années qu'on le constate, l'égalité et la parité ne sont pas automatiques. Comme cela a été rappelé tout au long de nos débats, malgré plusieurs lois sur ce sujet, les femmes restent victimes de discriminations et d'inégalités dans la sphère professionnelle. Des pénalités financières à hauteur de 1 % existent déjà, par exemple en cas d'absence d'accord sur l'égalité. On a désormais assez de recul, madame la rapporteure, pour conclure qu'elles ne sont pas assez dissuasives Pour les instances dirigeantes, fixer ces sanctions à 10 %, au maximum, des rémunérations et des gains aurait certainement un effet beaucoup plus persuasif.

diverses, souhaitaient que la sanction financière ne s'applique que sur le périmètre de la population concernée par la non-application des quotas.

elles n'embaucheront pas de femmes. Nous ne voulons absolument pas en arriver à une situation où les femmes seraient davantage discriminées

Seront ainsi soumises à l'obligation de quota les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif, ont employé un nombre moyen de plus de 1 000 salariés. En apportant cette précision, il s'agit d'éviter qu'une société qui franchirait ce seuil de façon temporaire ne sache pas si elle doit se conformer ou non aux obligations qui figurent à l'article 7. Cette formulation reprend, encore une fois, les modalités de la loi Copé-Zimmermann.

accélérer la mise en application des nouvelles dispositions instaurant des quotas pour les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes des entreprises d'au moins 1 000 salariés. 1 000 salariés. Dans sa version actuelle, l'article 7 prévoit l'application d'un quota de 30 % en 2027 et de 40 % en 2030, en laissant à chaque fois deux ans aux entreprises pour se mettre en conformité avec ces objectifs. Ces dispositions ne s'appliqueraient donc qu'en

dans certains bassins d'emploi, la parité est particulièrement déséquilibrée. La mesure que vous proposez reviendrait à faire évoluer de manière précipitée le corps social de l'entreprise, sans prendre en considération le déroulement des parcours professionnels déjà engagés

je trouve même que les femmes sont incroyablement patientes ! Qui d'autre que les femmes pourraient supporter autant d'inégalités

ne bloquent que rarement les ronds-points ou les péages d'autoroute, alors qu'elles auraient mille et une raisons de le faire. Elles sont très patientes

du Gouvernement ? Monsieur le sénateur, vous nous proposez de prévoir qu'une instance dirigeante puisse être mise en place non seulement au sein d'une société, mais également entre des sociétés comprises dans un même périmètre de consolidation au sens de l'article L.

Je suis favorable à cet amendement.

est à Mme Annick Billon. Le rapport d'information de la délégation aux droits des femmes du Sénat sur le bilan de l'application de la loi Copé-Zimmermann, laquelle a introduit des quotas de représentation de chaque sexe au sein des instances de gouvernance des entreprises, a montré que celui-ci était très positif dans les grandes sociétés cotées, mais que la mixité restait limitée dans les conseils d'administration et de surveillance des plus petites capitalisations boursières. Le présent amendement vise donc à affirmer le rôle des comités spécialisés spécialisés dans le respect de l'obligation de représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du conseil d'administration, ainsi que leur mission d'identification des profils dans les plans de succession des dirigeants mandataires sociaux. Il tend également à fixer des règles de représentation de chaque sexe au sein de ces comités, lesquels devraient

à Mme Martine Filleul. L'existence d'un vivier de femmes compétentes pour siéger dans les instances dirigeantes n'est plus à prouver aujourd'hui, mais elle amène à se poser la question de la limite du cumul des mandats dans les conseils d'administration. Limiter le nombre de mandats successifs à trois, contre cinq actuellement, libérerait des places dans les conseils et permettrait à davantage de femmes d'accéder à cette fonction.

Nous proposons donc de traduire cette proposition dans un amendement et de limiter le nombre de mandats d'administrateur pouvant être simultanément exercés par une même personne, afin de favoriser le renouvellement et, par là même, la parité dans les conseils d'administration.

? Ces deux amendements tendent à limiter à trois, au lieu de cinq actuellement, le nombre de mandats d'administrateur pouvant être cumulés par une même personne au sein des conseils d'administration.

madame la présidente, cette demande, pour surprenante qu'elle soit, a été largement soutenue par des instances éminemment importantes pour les entreprises.

en instituant une obligation pour les entreprises visées, sociétés anonymes et sociétés en commandite par actions de 250 salariés et plus, et présentant un chiffre d'affaires net de 50 millions d'euros et plus, ou un total de bilan d'au moins 50 millions d'euros, de déclarer annuellement au greffe du tribunal de commerce, soit annexée au registre du commerce et des sociétés, la composition de leurs organes de gouvernance ainsi que la répartition entre les femmes et les hommes au sein de chacun d'entre eux. Par ailleurs, cet amendement tend à faire de la composition des organes de gouvernance et de la répartition entre les femmes et les hommes au sein de ceux-ci une information obligatoire du rapport de gestion, afin d'en faciliter le contrôle. Enfin, les greffes des tribunaux de commerce sont tenus de vérifier l'obligation de dépôt et de mise à jour annuelle, le défaut d'information et de déclaration au registre du commerce et des sociétés étant susceptible d'une mise en demeure assortie d'une astreinte prononcée par le président de la juridiction commerciale. En tout état de cause, les dispositions prévues par le présent article sont de nature à responsabiliser les entreprises. Dans les sociétés dotées d'un commissaire aux comptes, celui-ci vérifie l'exactitude et la sincérité des informations transmises. Dans les autres sociétés, l'obligation déclarative, la publication de l'information et l'éventualité d'une mise en demeure assortie d'une astreinte mobilisent en amont les conseils de l'entreprise, au premier rang desquels les experts-comptables.

auteurs de cet amendement est louable, puisqu'il s'agit de renforcer la transparence concernant les obligations paritaires des entreprises. Cependant, le dispositif tel qu'il est proposé met sur le même plan les obligations issues de la loi Copé-Zimmermann et celles qui figurent

à Mme Laurence Cohen. Cet amendement vise à rétablir la rédaction issue de l'Assemblée nationale qui prévoyait la création d'un outil de contrôle intégrant la délibération annuelle des conseils d'administration et des conseils de surveillance, afin de mesurer les écarts de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes. est l'avis de la commission ? L'article 7 a été supprimé par la commission parce qu'il était superfétatoire. En effet, l'article 7 prévoit déjà que les données relatives à la répartition par sexe des cadres dirigeants et des membres des instances dirigeantes figurent au sein des bases de données économiques, sociales et environnementales. Les indicateurs qui y sont mentionnés sont pris en compte pour la délibération annuelle des organes d'administration sur la politique mise en oeuvre par la société en matière d'égalité professionnelle et salariale.

Le taux de rejet de crédits demandés par des créatrices d'entreprises est de 4,3 %, alors qu'il n'est que de 2,3 % pour les hommes. Les femmes sont ainsi près de deux fois plus nombreuses à essuyer des refus de prêts.

leur accès aux prêts. En conséquence, cet amendement travaillé avec la Fondation des Femmes vise à ce que Bpifrance fixe un objectif de mixité dans l'attribution des aides aux entrepreneurs et dans la facilitation de l'accès aux prêts.

Monge. Cet amendement a pour objet de supprimer le report à 2025 de la conditionnalité des prêts de Bpifrance et de la féminisation des comités d'investissement, introduit par la commission des affaires sociales du Sénat. En effet, il convient que les entreprises concernées s'approprient au plus tôt l'obligation de publication de l'index. Aussi, il ne nous semble pas justifié de reporter la conditionnalité de l'octroi de financements en fonds propres par la Banque publique d'investissement

pour que la situation évolue. Afin que les difficultés particulières rencontrées par les femmes entrepreneures soient mieux prises en compte, le présent amendement

Il s'agit de répondre aux alertes qui ont été précédemment portées au sein de notre assemblée. Ce rapport s'attacherait à présenter les modalités de mise en oeuvre de cette obligation, dans tous les territoires et à tous les niveaux de scolarité,

il est essentiel que le temps consacré à l'enseignement moral et civique soit l'occasion d'aborder également les questions relatives au respect de la dignité humaine et à l'égalité entre les femmes et les hommes. Cet amendement vise à insérer un alinéa en ce sens dans le code de l'éducation. Quel

fait acquérir aux élèves le respect de la personne, de ses origines et de ses différences, de l'égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que de la laïcité. La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut,

Les mesures visant à la mixité des formations, à une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, à la création de quotas permettant l'accès des femmes à des postes de direction doivent contribuer à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans la société. Ce texte permet également de lutter contre un certain sexisme financier qui limite l'accès des femmes aux financements pour le développement de leur entreprise. Le Sénat a su préserver les équilibres trouvés en favorisant l'accès des femmes à l'emploi, à l'entrepreneuriat et aux postes de direction, tout en évitant d'imposer de trop lourdes contraintes aux entreprises.